L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2020

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous nous retrouvons cet après-midi en séance pour la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire (CMP) sur le quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2020 le dernier, semble-t-il. Encore une fois, le calendrier a été particulièrement resserré, puisque, la semaine dernière, nous avons examiné ce texte en première lecture et, le lendemain, avons retrouvé nos collègues députés dans le cadre de la CMP. À l'occasion de À l'occasion de la première lecture, nous avons pris acte du fait que le Gouvernement a dû revoir à la baisse sa prévision de croissance pour 2020, avec une chute de 11 Ce scénario de croissance repose sur l'hypothèse d'une perte d'activité de 20 % par rapport au niveau d'avant-crise en novembre, contre 30 % en avril, lors du premier confinement.

la prévision de croissance gouvernementale inclut déjà une prolongation du confinement en décembre. De ce fait, c'est uniquement la hausse des dépenses liées aux mesures de soutien qui explique la dégradation de la trajectoire budgétaire dans ce texte. Comme vous le savez, ce renforcement porte prioritairement sur les mesures permettant de compenser directement les pertes des entreprises, avec le fonds de solidarité, les exonérations de cotisations sociales ou encore l'activité partielle. Le Gouvernement a donc fait le choix de la prudence. Le budget rectificatif repose sur des hypothèses extrêmement conservatoires, et le déficit annoncé ne devrait pas réellement être atteint. Des crédits budgétaires seront reportés sur 2021. Cela nous a déjà été confirmé dans le cadre de l'examen du PLF 2021, avec même l'ouverture de crédits complémentaires. Au total, les ouvertures de crédits au fil des quatre lois de finances rectificatives de 2020 sont dix fois plus élevées que les années précédentes. C'est, d'une certaine manière, colossal, mais c'est nécessaire. C'est la raison pour laquelle nous avons voté les trois précédentes lois de finances rectificatives et que nous voterons la quatrième aujourd'hui sans en modifier l'équilibre global. Les mesures de soutien sont là et bien dotées. Le Gouvernement garde indéniablement des marges de manoeuvre pour affronter les prochaines semaines et reste très prudent. La situation peut l'expliquer, mais nous veillerons à contrôler leur usage. Pour autant, le Sénat a procédé à quelques modifications, ajouts et suppressions qui répondaient à des attentes légitimes. Le travail de compromis que j'ai réalisé avec le rapporteur général de l'Assemblée nationale, Laurent Saint-Martin, a permis de reprendre plusieurs des apports significatifs du Sénat. Tout d'abord, nous avons préservé les crédits dédiés au sport, qui devaient initialement être annulés, à hauteur de 4,7 millions d'euros, ainsi que la suppression du rétablissement du droit à l'image collective. Pour autant, il nous faut soutenir le milieu sportif touché par la crise. De même, les crédits de la mission interministérielle de coordination anti-fraude (Micaf), qui subissait une annulation de 500 000 euros, ont été maintenus. Ensuite, afin de répondre aux préoccupations de notre assemblée, des crédits supplémentaires ont été votés, à raison, par exemple, de 20 millions d'euros à destination des Alpes-Maritimes, département durement touché par une tempête cet automne. 8 millions d'euros ont également été dégagés pour soutenir la filière équine dans la période de crise sanitaire et pour tenir compte des difficultés particulières auxquelles elle doit faire face.

Enfin, concernant les avances remboursables faites aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) pour compenser leurs pertes de recettes, la proposition du Sénat a été retenue. Celle-ci prévoit une clause de « retour à meilleure fortune selon laquelle ces autorités ne seraient tenues au remboursement des avances perçues qu'à compter de l'année suivant le retour d'un niveau de recettes équivalent aux années 2017 à 2019. Le principe d'un remboursement échelonné sur une période minimale de six ans a également été conservé. Certaines de nos autres propositions n'ont certes pas été conservées, mais des engagements ont été pris avec Laurent Saint-Martin pour que plusieurs dossiers avancent au cours des prochains mois. Ainsi en est-il, par exemple, du sujet de compensations des collectivités territoriales, sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure, lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances. Il conviendra de continuer de suivre avec attention les compensations aux collectivités territoriales pour couvrir les pertes de recettes subies. Par ailleurs, je considère que nous devons convaincre le Gouvernement de la nécessité de trouver un meilleur fonctionnement du fonds de solidarité, en particulier à l'égard des travailleurs indépendants. Nous avons été saisis de cas concrets qui montrent qu'un certain nombre d'acteurs économiques, commerçants, travailleurs indépendants et petits entrepreneurs, ne sont pas soutenus ou ne le sont pas Nous en sommes arrivés à la conclusion qu'il convient de prévoir, au-delà de l'aide de 1 500 euros, un renforcement du fonds de solidarité à leur profit, afin de tenir compte des charges fixes de ces structures. L'ensemble du tissu économique français doit être préservé. Je présenterai d'ailleurs un nouvel amendement sur le sujet dans le cadre de l'examen de la mission « Plan de relance » du PLF pour 2021. Pour conclure, je me félicite des avancées issues des travaux du Sénat auxquelles nous sommes parvenus sur ce quatrième projet de loi de finances rectificative, lequel s'inscrit dans la continuité des trois précédents textes que nous avons examinés. Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter les conclusions de la CMP, texte de compromis avec nos collègues députés. Cela ne nous empêchera pas de montrer les failles de votre politique, en particulier dans les choix que vous opérez pour la relance, monsieur le ministre.

Madame la présidente, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la dernière étape du quatrième projet de loi de finances rectificative pour 2020, à la suite de l'accord conclu en commission mixte paritaire. Depuis le début de la crise, les rectifications du budget pour 2020 ont abouti quatre fois à un accord entre les deux chambres. J'y vois le signe de l'esprit de responsabilité qui anime le Parlement depuis le début de cette crise. Je tiens à remercier l'ensemble des parlementaires pour leurs contributions, qui ont permis d'enrichir le débat et de préciser des points importants. Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, ce quatrième budget rectificatif pour 2020 a un double objectif : consolider les dispositifs de soutien ; ouvrir ou annuler les crédits dans le cadre du schéma de fin de gestion.

les débats, porté la volonté de renforcer l'ensemble des mesures de soutien à destination des secteurs touchés par les restrictions d'activité. Ces dispositifs seront poursuivis et dotés de nouveaux moyens. Ainsi, le fonds de solidarité sera rechargé de 10,9 milliards d'euros. L'activité partielle sera prolongée, ce qui portera son montant total à 34 milliards d'euros. Les exonérations de cotisations sociales atteindront 8,2 milliards d'euros, avec un réabondement, au total, de 4,3 milliards d'euros. De plus, une aide sera apportée aux personnes les plus vulnérables, avec le financement d'une prime exceptionnelle de 150 euros pour les allocataires de minima sociaux, logement (APL) et les étudiants boursiers, soit un accompagnement de 1,1 milliard d'euros. L'Assemblée nationale a, en outre, renforcé les aides destinées aux personnes les plus précaires par une dotation de 330 millions d'euros en autorisations d'engagement et 176,5 millions d'euros en crédits de paiement sur la mission « Travail et emploi ». Ces moyens supplémentaires permettront de créer 30 000 nouveaux postes dans le secteur de l'insertion par l'activité économique, mais aussi de développer l'emploi dans les quartiers prioritaires. Ils permettront également de financer le service public de l'insertion et de l'emploi. C'est un geste important pour renforcer l'accès au marché de l'emploi de ceux qui en sont le plus éloignés. Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à financer un nouveau dispositif d'urgence pour préserver l'emploi associatif, puisque nous savons que la crise sanitaire et économique a fragilisé le tissu des petites associations employeuses. La seconde vague épidémique et les mesures de restriction sanitaire qui les confrontent à de nouvelles difficultés et, parfois, menacent leur maintien nécessitent cette intervention. Cette mesure de soutien exceptionnel contribuera à préserver les emplois de plus de 5 000 petites associations touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire. L'examen de ce texte dans l'hémicycle du Sénat a permis d'élargir certaines mesures de soutien. Je fais référence notamment au vote de l'amendement de la commission des finances visant à étaler le remboursement des avances en faveur des autorités organisatrices de la mobilité sur une période minimale de six ans. Cet échelonnement permet de préserver les collectivités, qui commenceront à rembourser une fois qu'elles auront retrouvé une situation financière soutenable. Ces avances remboursables permettront, à court terme, de compenser les pertes de versement mobilité et de recettes tarifaires en région comme en Île-de-France, à hauteur de 1,95 milliard d'euros au total.

De plus, après l'adoption d'un amendement du Gouvernement, la mission « Enseignement scolaire » bénéficiera de 25 millions d'euros de crédits additionnels pour financer le recrutement d'assistants d'éducation dans les collèges et les lycées professionnels, afin de permettre aux enseignants vulnérables de dispenser leurs cours à distance tout en maintenant un encadrement des élèves dans les établissements. réunie la semaine dernière a confirmé l'ensemble de ces moyens supplémentaires. Je m'en félicite. En somme, les députés et sénateurs se sont accordés sur plusieurs points majeurs. Je tiens à saluer de nouveau la qualité de leurs travaux. Au-delà des dispositifs que je viens d'évoquer, je souhaite moi aussi mentionner l'allocation d'un soutien supplémentaire de 20 millions d'euros au département des Alpes-Maritimes, dans le cadre de l'effort de reconstruction consécutif au passage de la tempête Alex, qui a fait des dégâts historiques. S'il n'en prend pas la forme, ce soutien est clairement inspiré d'un amendement adopté par votre chambre. Par ailleurs, 8 millions d'euros ont été ouverts pour soutenir le secteur des centres équestres et poneys-clubs, en conformité avec les attentes de plusieurs parlementaires et en complément des aides débloquées au début de l'été. Enfin- c'est un sujet qui a fait l'objet de débats entre les deux chambres compte tenu de ses limites, le dispositif du droit à l'image collective applicable entre 2004 et 2010 ne sera pas réintroduit. Le Parlement a suivi, en cela, l'avis du Gouvernement et des rapporteurs généraux. Je veux de nouveau vous en remercier. Ce quatrième projet de budget rectificatif, bien qu'inédit, est en conformité avec les engagements du Gouvernement de ne pas inclure de nouvelles mesures fiscales pour l'année 2020. De plus, hormis les crédits d'urgence, il prévoit des ouvertures de crédits égales aux annulations, permettant ainsi un maintien du niveau révisé des crédits ouverts dans les différentes lois de finances rectificatives de cette année. Je veux terminer par deux remarques. Premièrement, je souscris aux propos de M. le rapporteur général concernant le travail qui reste à faire, notamment en matière de soutien aux travailleurs indépendants. Bruno Le Maire et moi-même travaillons actuellement à des dispositifs pour accompagner la sortie du

le texte. L'Assemblée nationale et le Sénat se sont accordés à quatre reprises sur les projets de loi de finances rectificative que nous avons présentés à votre examen au cours de la crise. Chaque fois, cela s'est fait dans un esprit de responsabilité. ce quatrième PLFR présente une particularité supplémentaire, qui est de porter le schéma de fin de gestion du PLF 2020, tel que voté initialement et tel que mis en oeuvre par le Gouvernement et sa majorité.

Ces trois accords, en avril, en juillet et en ce mois de novembre, ont, en outre, été précédés d'une adoption conforme du tout premier PLFR de 2020, en mars dernier, alors que la France voyait arriver la première vague épidémique. Nous pouvons tous nous en féliciter. À cet égard, monsieur le ministre, vous avez bien fait de saluer, à deux reprises, l'esprit de responsabilité du Sénat. Alors que le Sénat examine actuellement la première partie du projet de loi de finances pour 2021, je ne m'attarderai pas sur le contexte macroéconomique et la situation des finances publiques. Je me contenterai de rappeler que nous enregistrons aujourd'hui un triste record pour notre pays la dette et le déficit publics n'auront jamais été aussi élevés. La dépense publique, qui avoisine quant à elle les deux tiers de la richesse nationale, atteint, en 2020, en France, un montant vertigineux. Mais je ne veux pas verser dans la polémique. Nous savons tous que ces réalités découlent directement des décisions lourdes que nous avons prises afin de limiter la propagation du virus. Espérons et faisons en sorte que nous pourrons bientôt tourner la page. En tout état de cause, je me réjouis que l'Assemblée nationale ait accepté plusieurs des améliorations que le Sénat a apportées au texte. En effet, la gravité de la situation commande l'esprit de compromis.

Je me réjouis de cette solidarité, qui renforce la cohésion des territoires. Je pense également au renforcement de certaines aides sectorielles. Ainsi, la filière équine a vu ses recettes baisser et ses dépenses augmenter pendant la crise, alors que, ne pouvant plus accueillir de public, elle continuait de prodiguer les soins d'entretien aux chevaux. De nombreux acteurs de nos territoires sont concernés par cette situation exceptionnelle, qui demandait des moyens exceptionnels. Je me réjouis donc que la CMP ait retenu la solution proposée par notre collègue Jean-Pierre Vogel sur ce sujet. Ce sont ainsi 8 millions d'euros de crédits supplémentaires qui seront mobilisés. Enfin, je me réjouis que l'Assemblée nationale ne soit pas revenue sur la décision de supprimer l'article 1 A, qui rétablissait le droit à l'image collective pour les sportifs professionnels. De fait, il ne s'agissait pas d'une mesure de PLFR, comme M. le rapporteur général l'a rappelé. Je souhaite saluer ici la décision courageuse de la commission.

sur un certain nombre de dispositifs mis en place dès le début de la crise : chômage partiel, prêts garantis, fonds de soutien, etc. De fait, ces dispositifs sont bénéfiques pour le maintien de notre économie, et nous les voterions sans difficulté

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le temps est compté. Quand nous nous sommes réunis mardi dernier pour la CMP sur ce dernier budget rectificatif, il y avait urgence- il y a toujours urgence ! Nous avons su mettre de côté nos désaccords pour apporter une réponse claire et rapide à la crise. Il était nécessaire d'aboutir à une CMP conclusive, pour les bénéficiaires des aides et des mesures qui ont été votées afin de faire face à la seconde vague, pour accompagner ceux qui ont été touchés par les nouvelles mesures de restriction, décidées pour faire face au regain de l'épidémie. Il y allait de notre responsabilité de parlementaires. Le Gouvernement nous a transmis dans des délais tout à fait exceptionnels un projet de loi ambitieux, clair et simple, couvrant de larges champs de notre économie et permettant de répondre à de nombreuses angoisses économiques et sanitaires que nous voyions émerger dans le pays. Nous l'avons adopté dans des délais tout aussi exceptionnels. Plus vite nous adopterons ce texte de consensus, plus vite la loi sera promulguée, plus vite elle pourra commencer à produire ses effets pour nos concitoyens. Rappelons-le, la situation d'urgence ne veut pas dire que nous avons mis de côté notre responsabilité de parlementaires. Nous avons adopté de nombreuses mesures, qui ont enrichi le texte proposé par le Gouvernement. Reconnaissons toutefois

par en oublier l'ampleur : 20 milliards d'euros, qui s'ajoutent aux 66 milliards d'euros déjà dépensés depuis le début de la crise. Parmi les onze articles qui nous étaient soumis, le Sénat en a d'ailleurs adopté sept conformes. reconnaissance des efforts du Gouvernement, qui veille toujours à améliorer le soutien et la qualité des réponses de l'État à la crise. Comme vous l'avez reconnu durant la CMP, monsieur le rapporteur général, les ouvertures de crédits votées tout au long de l'année dans ces quatre budgets rectificatifs sont colossales, colossales, mais nécessaires. C'est pour cette raison que le Sénat a pris ses responsabilités et voté ces quatre textes. Je tiens, à cette occasion, à saluer l'attitude constructive de la majorité sénatoriale. Le Sénat a fait adopter plusieurs mesures dont le groupe RDPI salue l'ambition et la cohérence et qui ont été maintenues dans le texte final : nous avons maintenu les crédits dédiés au sport, dégagé 8 millions d'euros supplémentaires pour la filière équine et alloué 20 millions d'euros au département des Alpes-Maritimes, durement frappé par des catastrophes naturelles. Le Sénat a également prévu une clause de retour à meilleure fortune et un délai minimal de remboursement de six ans pour les avances aux autorités organisatrices de la mobilité. Ce sont elles aussi des mesures de bon sens,

n'était sans doute pas une réponse appropriée, et la CMP a voté en responsabilité pour sa suppression. Laurent Saint-Martin, rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale, a souhaité engager au plus vite une discussion avec le Gouvernement pour renforcer le soutien à ce secteur. le soutien à ce secteur. Je salue cet effort, qui doit intervenir le plus rapidement possible pour sauver ce qui peut être sauvé. C'est la logique d'un plan de soutien dans l'urgence. Une nouvelle fois, les parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat ont été au rendez-vous et à la hauteur des enjeux.

Entre son dépôt, le 4 novembre dernier à l'Assemblée nationale, et l'examen, aujourd'hui, de ses conclusions se seront écoulées trois courtes semaines, déjà bien occupées par le début de la discussion du PLF et par d'autres textes importants. Malgré cela, le nombre d'amendements en première lecture aura été relativement important, pour des sujets qui parfois relevaient davantage de 2021 paritaire est néanmoins parvenue à un accord, ce qui est un bon signe envoyé à nos concitoyens, dont certains ont besoin que les mesures contenues dans ce texte entrent en vigueur le plus rapidement possible. Si la situation sanitaire semble s'être légèrement améliorée par rapport à la semaine dernière, cette évolution est très progressive, irrégulière et incertaine au regard des risques de réémergence à tout moment de foyers épidémiques. L'exécutif réserve probablement ses principales annonces pour l'allocution de ce soir Le Gouvernement peut-il néanmoins d'ores et déjà suggérer quelques orientations ? On l'a dit : la chute de l'activité lors du premier confinement a été complètement inédite depuis au moins la dernière guerre. L'activité a toutefois connu, pendant l'été, mais dont on sait désormais que le prix à payer sont les mesures de reconfinement et les nouvelles restrictions de cet automne. Nous ne sous-estimons pas la gravité de la situation : la tentation est

Force est de constater, jusqu'à présent, de véritables difficultés dans la capacité à contrôler cette situation sanitaire et à en limiter les effets sur le reste de la sphère sociale.

de ce sombre diagnostic, il faut saluer les mesures contenues dans ce PLFR, et le consensus auquel sont parvenus les parlementaires des deux chambres. Si des déceptions existent- je citerai la non-prise en compte de certains secteurs comme celui des loisirs,

Le temps viendra de faire les comptes de cette année en tous points exceptionnelle et de veiller, en particulier, à la résorption de l'endettement, désormais colossal. De ce point de vue, les négociations actuellement en cours à Bruxelles entre partenaires européens sont décisives ; comme souvent, elles sont un test de la résistance de la communauté européenne en période de crise. Voilà les quelques remarques que je souhaitais formuler sur ces conclusions

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans les quatre minutes qui nous sont imparties, nous ferons quelques observations rapides sur les données de ce quatrième collectif budgétaire de l'année, dont le moins que l'on puisse dire est que les modifications qu'il contient ne sont, au fond, que très marginales. Pour autant, notons tout d'abord que les membres de la CMP ont pu se mettre d'accord sur un texte commun, qui consiste à supprimer beaucoup des apports de la première partie. J'en veux pour exemple l'amendement visant à créer une taxe sur les services numériques, qui, une nouvelle fois, est passé à la moulinette de la CMP. Adopté pour la troisième fois dans cet hémicycle il y a encore quelques jours, dans le PLF en cours d'examen, son vote définitif permettrait de faire contribuer les acteurs du numérique au plus proche du niveau de leurs activités réelles sur le territoire français. Il renforcerait la taxe sur les services numériques dite « GAFA », que d'aucuns considèrent comme largement insuffisante, et pallierait l'impunité de ces entreprises qui ne connaissent pas la crise économique. Le déficit s'envole pour soutenir les entreprises, soit, mais ne profite nullement à la demande.

150 euros : autrement dit, 220 milliards d'euros pour les entreprises, 1,1 milliard pour les plus démunis, le jour même de l'ouverture des Restos du coeur et à l'avant-veille de la publication du rapport de l'Observatoire des inégalités, comme si urgence économique et urgence sociale ne devaient pas aller de pair ; comme si aider massivement les entreprises à passer la crise sanitaire pouvait suffire à résoudre la crise sociale, qui est déjà bien présente comme si l'une n'était pas fonction de l'autre ! Je ne peux ici que constater, entre nous, une divergence profonde et manifeste. Nos débats semblent parfois, voire trop souvent, complètement déconnectés de ce que nos concitoyens et concitoyennes vivent dans cette période très exceptionnelle. De mars à fin septembre, l'État a ainsi engagé 25 milliards d'euros dans le plan d'urgence, dont 22 ont été accordés aux entreprises, notamment pour financer l'activité partielle. Celle-ci a au tiers été supportée par l'Unédic, par le biais de sa dette garantie par l'État, tandis que la sécurité sociale a dû consentir à plus de 44 milliards d'euros d'exonérations totales ou de reports de cotisations. Parallèlement, les collectivités locales, elles, n'ont pu que constater des pertes de recettes non totalement compensées. est des prêts garantis par l'État, ils partirent 300 mais arrivèrent 120- je parle en milliards d'euros -, permettant aux banques de transformer des crédits de court terme en prêts de moyen voire de long terme, plus juteux en intérêts encourus Vous avez négocié les taux d'intérêt, mais ils peuvent tout de même atteindre 2,5 %. Parmi les entreprises concernées, nombres d'entre elles, quoi qu'on en ait dit, n'ont pu se voir prêter la somme qu'elles avaient demandée. pour le reste, comme à l'accoutumée : ouverture de crédits pour compenser les insuffisances initiales, notamment en matière d'action sociale de l'État- mais c'est là une habitude ancienne. La vérité est que ce collectif tourne le dos aux maux qui minent notre société et notre économie. Il aura suffi d'un terrible virus pour supprimer plus de 800 000 emplois dans ce pays et révéler, en quelques jours,

les politiques de « maîtrise des dépenses publiques » ont privé notre pays, puissance économique de référence dans le monde en matière de santé publique, de sa capacité d'agir en prévention comme en réparation.

soit fait pour identifier les difficultés. Disons-le clairement : pour ce qui est des moyens mobilisés pour apporter des compensations aux différents acteurs économiques, il manque encore des choses

ce fonds de solidarité apporte un certain nombre de réponses aux besoins des acteurs économiques ; je pense bien sûr aux commerçants dont les activités ne peuvent se poursuivre, aux indépendants qui ne sont pas toujours aidés comme il le

ils ne fonctionnent plus. Mais ils n'ont droit à aucune compensation, si ce n'est, bien sûr, pour leurs salariés, le recours à l'activité partielle. Comment voulez-vous qu'ils fassent face aux charges qu'ils ont à assumer ? C'est tout

égard : un effort réel a été consenti -, mais il importe que l'on prenne en compte la réalité des situations identifiées sur les territoires ; or tel n'est pas encore le cas. Il reste beaucoup à faire et il est

que les activités économiques qui aujourd'hui ne peuvent fonctionner puissent enfin reprendre, avec- je l'ai dit -les précautions sanitaires qui s'imposent. Nous souhaitons aussi que nos concitoyens puissent avoir un peu plus de liberté de circulation. Disons-le sans

Féraud. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est sans surprise que la commission mixte paritaire sur ce projet de loi de finances rectificative a été conclusive. Sur la forme, nous pourrions bien sûr nous montrer satisfaits que nos deux assemblées s'entendent sur un texte aussi important dans la période de violente crise économique et sociale que nous traversons, cet accord le rendant applicable rapidement. Malheureusement, nous ne pouvons pas nous en contenter, tant le texte issu des travaux de la CMP est proche du projet de loi initial du Gouvernement, et tant nos inquiétudes sur le sort des plus précaires de nos concitoyens restent fortes à l'issue de la discussion parlementaire. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera donc de nouveau contre. Sur le fond, en effet, qu'est-ce qui a changé dans ce PLFR 4 ? Rien ou presque, puisque la majorité sénatoriale a elle-même accepté de reporter l'introduction de toute nouvelle mesure importante à l'examen du projet de loi de finances. Avec les sénatrices et sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, nous avions obtenu deux avancées lors de la discussion de ce PLFR en première lecture : premièrement, le déplafonnement du montant de la compensation versée par l'État aux autorités organisatrices de la mobilité, pour un montant d'environ 45 millions d'euros, sur l'initiative de notre collègue Olivier Jacquin

Mais ces deux avancées votées par le Sénat ont été supprimées du texte, au motif- ce motif était un engagement, toujours le même -que nous y reviendrions au cours de l'examen du PLF. Nous verrons bien si tel sera le cas, et nous saurons, monsieur le

bien été rétablis. Nous avons obtenu un fonds de soutien au département des Alpes-Maritimes à la suite des dramatiques inondations des dernières semaines, ou encore la mise sous garantie de retour à meilleure fortune des avances remboursables faites aux autorités organisatrice

Il aurait fallu des mesures choc pour permettre enfin aux Français les plus modestes comme aux entreprises les plus affectées de surmonter cette crise Il aurait fallu prendre à bras-le-corps l'enjeu de la pauvreté et soutenir beaucoup plus massivement la jeunesse. Il aurait fallu faire de l'urgence sociale une priorité politique.

montre que le Gouvernement ne semble pas beaucoup plus enclin à accepter nos propositions en faveur des victimes de la crise dans ledit PLF qu'il ne l'était lors de la discussion de ce projet de loi de finances rectificative. Pour toutes

triste et regrettable série d'une année qui aura profondément bouleversé nos vies sur le plan sanitaire, évidemment, mais aussi, de manière plus profonde, sur le plan économique. L'année 2020 est l'année des stupéfactions. Stupéfaction, d'abord, face à un virus méconnu arrivé sur notre territoire il y a près d'un an : il a poussé notre pays à s'enfermer, à s'isoler, à opter pour ce que nous n'avions jamais connu. Stupéfaction, ensuite, sur le plan économique : trois mois durant, ce sont des entreprises de toute taille qui ont souffert, parfois jusqu'à en mourir, n'ayant plus les rentrées d'argent ou la trésorerie nécessaires pour pouvoir honorer leurs charges. Stupéfaction, enfin, quant à l'attitude de votre gouvernement : sans consultation ni concertation avec le Parlement et avec les parties prenantes, vous avez décidé de renouer avec la même politique d'arrêt de notre économie qui avait déjà tant coûté à nos entreprises quelques mois plus tôt. Pourtant, dès le mois de mars, malgré la mise à l'écart du Parlement, devenue habituelle, dans la prise de décision du Gouvernement, nous vous alertions et acceptions de faire front commun face à cette crise en souscrivant aux mesures d'aide d'urgence destinées à préserver nos entreprises et nos emplois. Le Sénat a voté les trois premiers projets de loi de finances rectificative par responsabilité, parce que la situation imposait la solidarité de toute la Nation. Dans ce même esprit de responsabilité, le Sénat a décidé, la semaine dernière, en commission mixte paritaire, d'adopter ce quatrième PLFR, dans une situation qui a pourtant bien changé depuis mars, et dont il faut évidemment redéfinir ensemble les contours avant le vote final. Vous sollicitez aujourd'hui le Parlement pour qu'il vous autorise à débloquer 20 milliards d'euros supplémentaires pour financer les commerces de proximité, ceux que vous qualifiez de « non essentiels », parce que vous avez fait le choix du confinement, alors même que toutes les études scientifiques ont démontré que ces commerces n'étaient pas des lieux de contamination. Fermer ces commerces sans fermer les métros, vous avouerez que, quand on a du bon sens, c'est à n'y rien comprendre Toutes ces mesures auraient pu être évitées, j'en suis persuadé ... En réalité, ces choix ont été pris sans concertation avec le Parlement, mais uniquement sous avis médical, sans en mesurer les conséquences économiques et humaines pour les Français Nous sommes tous, parlementaires comme maires, confrontés à des chefs d'entreprise ou à des indépendants qui aujourd'hui n'en peuvent plus, et ne pensent pas pouvoir se relever de la situation dramatique dans laquelle vous les avez plongés. Beaucoup d'entre eux sont exténués et découragés, et ne savent plus comment faire pour éviter la mise en liquidation de leur entreprise. Ce confinement qui appelle un nouveau projet de loi de finances rectificative est un désastre, et les Français ne comprennent pas son manque de cohérence.

Le résultat de votre politique, en effet, c'est que toutes les entreprises du secteur tertiaire qui concourent massivement à la richesse de l'État sont aujourd'hui à l'arrêt ; et ce sont les Gafam, que vous n'êtes pas parvenus à taxer, qui en perçoivent la majorité des bénéfices. Vous revenez une quatrième fois devant nous pour vous aider à financer les échecs de vos choix et nous demander une énième autorisation de débloquer des aides pour les entreprises. Si, évidemment, nous le faisons, c'est parce que nous n'avons pas le choix. le choix. Les entreprises en ont besoin ; elles ne sont pas responsables de la situation dans laquelle elles se trouvent. Mais nous attendons de votre part de la sincérité. Monsieur le ministre, les Français veulent un discours de vérité sur le devenir des finances de notre pays. D'un côté vous diminuez les recettes de l'État, de l'autre vous continuez d'augmenter les dépenses, contrairement à vos engagements de campagne- je tiens à le répéter -et parce que vous êtes incapable de réformer. Bilan : par facilité, vous avez recours à la dette, cette dette qui est de moins en moins souveraine et qui, un jour, si les taux d'intérêt augmentent, deviendra insoutenable ! La Chine, aujourd'hui, prête à taux négatif : pensez-vous qu'elle le fasse par bonté ? Pour ma part, j'en doute un peu ... Quel avenir assurons-nous à nos enfants ? Votre espoir repose sur la croissance, mais combien d'années faudra-t-il pour retrouver le niveau de 2019 ? Et êtes-vous réellement convaincus que votre plan sera la solution, alors que nous ne sommes même pas capables de calculer la valeur ajoutée des investissements qui sont choisis ? Et que dire de cette idée folle du non-remboursement de la dette ? Faites-vous partie de ces analystes qui y croient ? Est-ce l'échéance de 2022 qui vous pousse à gérer ainsi ? Il est irresponsable de voter cette dérive financière ; en même temps, si nous ne le faisons pas, nous sacrifions tous les indépendants qui attendent ces ressources pour vivre

Les Français nous ont fait confiance, et j'ai de plus en plus le sentiment de les tromper, car nous n'arrivons pas à stopper la machine infernale du recours à la dette. Ce PLFR 4 nous amène à un point de non-retour, celui des presque 65 % de dépense publique, d'un déficit public creusé

du PLF 2021. Ce PLF doit être l'occasion pour vous de nous présenter un budget sincère en prenant en compte les préoccupations des Français et en vous fiant aux propositions et à la vision du Sénat notamment.

Nous le faisons pour nos entreprises et pour nos emplois, mais nous vous demandons solennellement d'arrêter de mettre de côté le Parlement dans l'élaboration de vos politiques, de permettre aux Français de travailler et de faire preuve de sincérité envers eux dans votre programmation budgétaire.

Le scrutin est ouvert.

est présenté par MM. Kern (TGAP) « amont ». Nous savons très bien qu'aujourd'hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs (REP), 50 % des déchets faisant l'objet d'un stockage ne bénéficient d'aucune filière de recyclage ni d'aucune filière de REP.

vers l'économie circulaire. C'est une sorte de prime au cancre ! Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable. Cet amendement vise donc à mettre en place une TGAP amont, envisagée à 0,03 euro par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la REP et ne pouvant faire la démonstration de l'existence d'une filière de récupération. Voilà

visent à mettre en place une nouvelle contribution, qui s'appliquerait à l'ensemble des « produits manufacturés » non couverts par une filière de responsabilité élargie du producteur.

notre peu d'entrain à la création de nouvelles taxes, quand bien même ce sujet est identifié comme problématique et devant faire l'objet d'un règlement dans les mois et les années à venir. La parole est

? Les réceptions de déchets dans des installations autorisées, mais ne respectant pas les prescriptions de ces autorisations, sont assujetties à un tarif majoré de TGAP. L'amendement vise à supprimer cette majoration pour les déchets reçus pendant la crise sanitaire. J'entends bien que les mois de confinement ont entraîné une mise à l'arrêt

malgré la crise sanitaire, et au regard des surcoûts auxquels le service public doit faire face, cet amendement vise à exonérer les collectivités de TGAP pour les déchets traités pendant la période d'état d'urgence sanitaire.

des efforts pourront peut-être être réalisés sur le coût d'exploitation, et donc sur les taxes ou redevances l'année prochaine. Mais il faut savoir que les structures qui portent ces installations

Ils sont donc nécessairement éliminés dans les installations de stockage et de traitement thermique. Les collectivités doivent payer la TGAP pour l'élimination de ces déchets. Pourtant, n'ont de prise ni sur la conception de ces produits, qui n'ont aucune filière de recyclage, ni sur leur mise sur le marché, ni sur leur consommation. Il semble donc injuste de les taxer pour l'élimination de ces déchets

franchise de TGAP déchets pour certains des déchets assimilés à des déchets ménagers pour les collectivités territoriales.

qui ne peuvent être recyclés et en permettant ainsi la production d'une énergie locale. Les unités de valorisation énergétique de CSR ne sont pas directement soumises à la TGAP sur les déchets réceptionnés en entrée. Toutefois, la TGAP reste applicable aux refus issus d'unités de préparation de CSR qui doivent être orientés en incinération ou en stockage. Une exonération de TGAP sur ces refus pourrait être un levier de développement de la filière.

l'amendement n° I-570. Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu'elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage. La nouvelle augmentation de la TGAP proposée par le Gouvernement fonctionnera de la même manière. Elle pénaliserait en premier lieu les collectivités, qui sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets. Cet amendement vise à compléter ce dispositif par un volet incitatif. Il créerait ainsi une réfaction de TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l'objectif de réduction du stockage porté par le Gouvernement, soit une division par deux des déchets envoyés en stockage par rapport à 2010. Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal en vigueur sur l'élimination des déchets, en maintenant un signal prix sur le stockage et l'incinération pour les collectivités qui n'ont pas atteint leurs objectifs de réduction du stockage, tout en évitant de sanctionner lourdement les collectivités qui ont réalisé les efforts.

Les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ont été fortement mobilisées pendant la crise sanitaire pour continuer à assurer la gestion des déchets des Français tout en garantissant la sécurité des agents et des usagers. Elles ont déployé des efforts considérables, qui ont été salués à juste titre par le Gouvernement, pour assurer ce service public essentiel dans des conditions difficiles. Cet amendement vise à reporter d'un an reporter d'un an l'augmentation de la TGAP issue de la loi de finances pour 2019. Cette mesure serait un acte de solidarité nationale.

De 9,15 euros la tonne en 2000, elle est actuellement de 17 euros la tonne, et elle s'élèvera à 30 euros en 2021. Cette hausse contraindra une nouvelle fois les collectivités territoriales à augmenter leurs tarifs aux usagers,

Ce report d'un an de la hausse de la TGAP permettrait aux collectivités territoriales de disposer des moyens nécessaires pour financer dans les prochaines années les dépenses qui s'imposent pour la mise en place de cette économie circulaire. Il permettrait également d'éviter que les collectivités soient sanctionnées financièrement en raison du retard pris par le Gouvernement sur la publication des textes d'application de la loi AGEC, ainsi que pour les mesures qui ont été rendues nécessaires par la crise sanitaire. Sans ce report, cette hausse serait répercutée sur le contribuable local, ce qui, dans le contexte actuel, fragiliserait encore davantage la population. Je vous remercie l'augmentation de la TGAP issue de la loi de finances pour 2019. Bien que la volonté de mettre un signal prix sur l'élimination des déchets pour favoriser le recyclage soit positive, cette réforme passe à côté de son objet et entraîne simplement une hausse des taxes payées par les collectivités pour la gestion des déchets, qui représentent 25 % du coût du service public. Dans le même temps, les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets ont été fortement mobilisées pendant la crise sanitaire pour continuer à assurer la gestion des déchets des Français tout en garantissant la sécurité des agents et des usagers. Elles ont déployé des efforts considérables, qui ont été salués à juste titre par le Gouvernement, pour assurer ce service public essentiel dans des conditions difficiles. Cette mesure serait un acte de solidarité nationale pour permettre aux collectivités de disposer des moyens nécessaires pour maintenir le cap du développement de l'économie circulaire, qui supposera d'importantes dépenses dans les années à venir. Elle permettrait également d'éviter que les collectivités soient sanctionnées financièrement en raison du retard pris par le Gouvernement sur la publication des textes d'application de la loi AGEC,

M. Didier Rambaud. Pour des raisons géographiques, démographiques et climatiques, les collectivités de Guyane et de Mayotte font face à d'importantes difficultés en matière de gestion des déchets, même si des efforts importants ont été accomplis pour mettre aux normes les installations de stockage. C'est pourquoi il est proposé de revoir la trajectoire d'augmentation des tarifs de la TGAP applicables à ces deux territoires, en prévoyant une réfaction de 75 % de 2021 à 2023, puis de 70 % à partir de 2024, contre 60 % actuellement. S'agissant des sites de stockage isolés guyanais, non accessibles par voie terrestre, ceux-ci avaient été jusqu'à présent pris en compte par la fixation d'une TGAP préférentielle à 3 euros la tonne. La situation de ces sites non accessibles par la route demeure très délicate et ne doit pas être aggravée par une augmentation de la TGAP. Le maintien d'un montant très bas à 3 euros par tonne est donc proposé pour ces sites.

Cette hausse de la TGAP n'a donc plus rien d'incitatif pour les DROM et les COM, qui font face à la réalité de la gestion des déchets en milieu insulaire. À titre d'exemple, à La Réunion, où sont enfouis tous les ans 380 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés, la TGAP pour les ménages coûtera 3,4 millions d'euros de plus en 2021, puis augmentera de 2 millions par an, pour atteindre 11,4 millions d'augmentation en 2025.

La population subira, de façon injuste, l'augmentation de cette taxe, faute d'équipements adaptés de valorisation des déchets, lesquels sont complexes à réaliser au vu des contraintes insulaires. Cet amendement vise donc à suspendre l'augmentation de la trajectoire de la TGAP dans les collectivités d'outre-mer à partir de 2021.

TGAP à La Réunion, en Guadeloupe, à la Martinique, mais aussi en Guyane et à Mayotte soit abaissé non plus de 60 %, mais de 75 %. Cette baisse passerait à 70 % en 2024.

Ainsi, de nombreuses installations de valorisation énergétique des déchets ont perdu des débouchés importants pour valoriser la chaleur fatale issue du traitement thermique. Dans ce contexte, il est possible que cette fermeture inattendue de débouchés pour la chaleur fatale entraîne une baisse du rendement énergétique, qui ferait passer certaines installations en deçà du seuil de 65 % permettant de bénéficier d'une réfaction de TGAP. Pour éviter que les collectivités et les opérateurs qui exploitent ces installations ne soient pénalisés fiscalement pour des événements qui ne relèvent pas de leurs actions, il est proposé d'assouplir le calcul du rendement énergétique pour l'année 2020.

Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal en vigueur sur l'élimination des déchets, en maintenant un signal prix fort sur le stockage et l'incinération pour les collectivités qui n'ont pas atteint leurs objectifs de réduction du stockage, tout en évitant de sanctionner lourdement les collectivités qui ont réalisé les efforts. Afin de simplifier la mise en oeuvre de cette réfaction, et notamment les difficultés liées à l'identification des tonnages issus des collectivités performantes, nous proposons d'instaurer cette réfaction sous forme d'un reversement des recettes de la TGAP aux collectivités ayant atteint leurs objectifs de stockage. Ainsi, les installations de traitement resteraient assujetties à la TGAP, et n'auraient pas à distinguer les taux à appliquer entre les différentes collectivités ou entreprises dont elles réceptionnent les déchets. En réduisant l'impact sur les finances publiques à 100 millions d'euros, cet amendement crée un effet incitatif très important pour les premières collectivités qui atteindront l'objectif de division par deux du stockage prévu par la loi de transition énergétique.

je le rappelle, est payée par les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu'elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage. Augmenter la taxe n'est pas suffisant pour modifier les pratiques. Puisque le Gouvernement souhaite augmenter la TGAP, il est indispensable d'envisager un mécanisme vertueux d'accompagnement. Tel est l'objet de cet amendement, qui prévoit d'instaurer une réfaction de la TGAP pour les collectivités qui sont parvenues à atteindre l'objectif, porté par le Gouvernement, Cela maintiendrait un fort signal prix sur les collectivités qui n'ont pas atteint leurs objectifs de réduction du stockage et récompenserait celles qui ont fait des efforts. L'objectif n'est pas de créer une usine à gaz incompréhensible, même si la gestion des déchets des usines à gaz est un sujet en soi

Je confirme à M. Mandelli que la subvention versée à l'Ademe baissera de 37 millions d'euros en 2021, par rapport à la dotation proposée en 2020.

-, une filière naissante, en subissent les conséquences. Il est aujourd'hui complexe pour eux de dégager des marges financières nécessaires à leur développement, à l'encaissement des coûts de recherche et d'homologation des véhicules. Cet amendement vise à soutenir la filière du rétrofit français, une filière d'excellence et d'avenir qui s'emploie à changer la motorisation de véhicules thermiques vers la traction électrique elle permet de donner une seconde vie plus vertueuse à des véhicules polluants sans les mettre au rebut ; elle rénove une partie du parc roulant sans avoir à construire de nouveaux véhicules ; elle permet une création de valeur, source d'emplois non délocalisables. C'est pourquoi les aides à l'acquisition de véhicules rétrofités doivent être consolidées. En mai dernier, le rétrofit de véhicules a été rendu éligible à la prime à la conversion. Mais il convient d'adapter le montant de la prime à la taille du véhicule. Cet amendement, porté par Nathalie Delattre,

des bateaux de ce calibre, l'ancien rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, Joël Giraud, notait dans son rapport sur l'application des mesures fiscales, en juillet 2019 : « Les explications pour le moins obscures de la douane ne permettent pas d'expliquer le rendement très décevant de cette mesure. »

Merci

Quel mauvais signal envoyez-vous ! Le pouvoir réchauffant de ces gaz est jusqu'à 15 000 fois supérieur à celui du CO2 ; ils ont des conséquences extrêmement néfastes et sont responsables de 5 % des gaz à effet de serre de la France. Même modeste, cette taxe a le mérite d'inciter à moins utiliser ce type de gaz très polluant et pousse les industriels à s'engager dans la transition énergétique.

L'article 16 prévoit de supprimer les prélèvements progressifs et complémentaires sur les casinos embarqués, au motif que leur rendement est nul. nul. Il n'explique pas en quoi l'objectif d'harmonisation fiscale, qui avait présidé à l'instauration de ces prélèvements dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2017, ne serait plus valide aujourd'hui. En outre, il maintient d'autres taxes pesant sur les mêmes casinos embarqués. Il est donc proposé de revenir sur cette volonté d'abrogation, dans l'attente d'un examen plus approfondi de la fiscalité de ces casinos. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pu disposer d'un état précis de la situation nous permettant, éventuellement,

Cette taxe frappe la réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires ainsi que les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à disposition du public. Le rendement de cette taxe ayant atteint

de marketing engagés par les entreprises, ainsi que sur le chiffre d'affaires des régies publicitaires. Sur 3 millions d'entreprises, moins de 1 % ont accès au marché publicitaire. En 2014, plus de 600 entreprises, soit 0,02 % d'entre elles, effectuaient

dont le développement problématique n'a été que temporairement freiné par la crise sanitaire. Ce taux de 25 % est volontairement important, car nous souhaitons désinciter fortement leur installation et limiter le recours à de tels panneaux pour les seuls cas où ils seraient vraiment nécessaires.

le consommateur, qui prime toujours. On regrette qu'il n'y ait plus de citoyens : il faut savoir ce que nous voulons ! Lorsqu'on crée du consommateur, on finit par n'avoir que du consommateur. Ces écrans numériques sont aussi une agression permanente dans la rue

25 euros sur les actes constatant des baux et sous-baux à durée limitée d'immeubles. Je tiens à faire observer que la formalité d'enregistrement n'est pas obligatoire pour ces actes. Le droit fixe n'est donc perçu que si les personnes concernées décident, volontairement, de les soumettre à l'enregistrement. En conséquence, il ne me paraît pas exagéré d'exiger le paiement du droit dans ce cas, puisqu'il est presque volontaire et souhaité. Je demande donc le retrait

avant cette taxe avait permis à l'État de collecter de nombreuses données sur le sous-sol profond, grâce aux activités d'exploration menées par les entreprises. Cette taxe est d'un rendement extrêmement faible de moins de 1 million d'euros : 810 000 euros en 2018 et une estimation de 50 000 euros pour 2022. Dès 2017, la commission des finances du Sénat a pu souligner que le rendement faible de la taxe était de nature à l'amener à disparaître d'ici une décennie quand l'ensemble des permis exclusifs de recherche sera arrivé en fin de validité. Les recettes ne permettront pas d'aider les collectivités à réaliser des projets de reconversion des territoires explorés.

en prie, ma chère collègue. Les HFC sont utilisés dans la réfrigération et dans la propulsion d'aérosols. Ils ont été mis en place pour remplacer les chlorofluorocarbures, les CFC, qui étaient responsables de la destruction de la couche d'ozone

est extrêmement important. Ce gaz figure parmi les six principaux gaz à effet de serre listés par le protocole de Kyoto, en 1997. Un accord mondial, conclu à Kigali en 2016, a fixé un calendrier

dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs. La réflexion n'a pas encore commencé et il me paraîtrait prématuré de supprimer ces taxes et de priver ainsi de plus de 250 millions d'euros de recettes en 2021. Pour aller au bout de ma réflexion, j'ai bien conscience que la SNCF enregistre des pertes très importantes en 2020, 4,7 milliards d'euros, dont 4 milliards sous forme de capitalisation, dans le cadre du plan de relance. La suppression de ces deux taxes

connaissons tous l'enjeu majeur de la lutte contre l'artificialisation des terres et l'étalement urbain, et nous savons également à quel point les grandes surfaces, les hypermarchés, sont des consommateurs de terres agricoles et des facteurs d'étalement urbain.

est de lever un frein important au recours à l'épargne en coopérative, dans le cadre de la dotation pour épargne de précaution (DEP). Cette modalité de constitution de l'épargne professionnelle permet à l'associé coopérateur de bénéficier, un contrat pluriannuel conclu avec sa coopérative, d'une plus grande stabilité des revenus qu'il tire de celle-ci. En effet, quand les prix de l'année sont au-dessus d'un prix de référence, l'exploitant ne reçoit que le prix de référence et la différence avec le prix de vente réel constitue une créance représentative de l'épargne de précaution. L'objet de cet amendement vise donc à permettre à l'exploitant de transférer, notamment dans l'hypothèse d'un retrait, retrait, le montant de ces créances sur le compte d'épargne monétaire en banque dédié à la DEP, à l'instar de ce que la loi prévoit pour l'épargne constituée sur des stocks en cas de vente de ces derniers. L'effort d'épargne ayant déjà été réalisé au niveau de la coopérative, il est incohérent d'y appliquer le plafond propre à la constitution d'une nouvelle déduction, puisqu'il s'agit non pas d'une nouvelle déduction, mais bien d'un transfert d'une épargne en créance en épargne monétaire.

donc à permettre à l'exploitant de transférer le montant de ces créances sur le compte d'épargne monétaire classique dédié à la DEP, à l'instar de ce que la loi prévoit pour l'épargne constituée sur des stocks en cas de vente de ces derniers. L'effort d'épargne ayant déjà été réalisé au niveau de la coopérative, il n'est pas très cohérent d'y appliquer le plafond propre à la constitution d'une nouvelle déduction, puisqu'il s'agit non pas d'une nouvelle déduction, mais bien d'un transfert d'une épargne en créance en épargne monétaire.

? Ces amendements visent à neutraliser les effets de la sortie d'une coopérative sur le sort de l'épargne constituée, à travers la constatation de créances sur la coopérative et par l'associé coopérateur au moment où il sort, au regard des règles

plusieurs actions tendent à diminuer la portée de la comptabilité et des informations publiques sur les entreprises, qui doivent permettre le contrôle efficace de leur action.

vise des actes clairement identifiés. Je ne suis pas sûr que la mobilisation des effectifs de l'administration fiscale sur des missions d'enregistrement des actes de société

en clair, d'ajouter une redevance additionnelle sur les sections d'autoroute soumises à péage. La directive 2011/76/UE du 27 septembre 2011 dite « Eurovignette 3 » permet en effet aux États membres d'introduire dans les péages routiers des poids lourds une prise en compte

En l'état actuel des choses- le passé nous le rappellerait utilement -, la création de cette taxe ne manquerait pas de provoquer

est à Mme Isabelle Briquet. Cet amendement vise à proroger de deux ans le dispositif de minoration de moitié des intérêts de retard applicables aux créances en matière d'impôts, de droits et de taxes, qui avait été introduit en loi de finances rectificative pour 2017. 2017. Au regard du contexte économique et social actuel, il paraît pertinent de maintenir ce dispositif pour deux ans, en attendant un rebond de l'économie, afin de ne pas amplifier les difficultés des contribuables, qui font actuellement les frais de la crise sanitaire, économique et sociale.

et prévenir ainsi les risques d'instabilité. En faisant cette proposition, l'économiste américain James Tobin, proposait dès 1968 de mettre un « grain de sable » dans les marchés financiers. Taxer un petit montant sur chaque transaction permet à la fois de générer des ressources pour l'État, mais aussi de tracer les mouvements de fonds pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale, et surtout de pénaliser les acteurs qui multiplient les petites opérations d'arbitrage ou de spéculation à des fréquences toujours croissantes, et qui contribuent largement à l'instabilité financière. Selon la proposition de l'association Attac, en taxant les transactions sur les actions et les produits structurés à 0,1 % et certains produits dérivés à 0,01 %, pourrions dégager 36 milliards d'euros par an à l'échelle européenne, dont 10,8 milliards d'euros pour la France. En comparaison, les recettes issues de la pseudo-TTF française, qui n'est en réalité qu'un simple impôt boursier, sont négligeables. négligeables. Le Président de la République n'a pas honoré sa promesse faite aux ONG de soutenir la mise en place rapide d'une TTF au niveau européen. Il incarne aujourd'hui l'un des principaux blocages face à la volonté du Parlement européen. En plus de la mise en place du dispositif que nous proposons, nous demandons donc, aux côtés des associations, notamment d'Attac, que la France soutienne le projet de TTF négocié par dix pays de l'Union européenne et que l'ensemble des transactions financières entre dans le périmètre de cette taxe. L'amendement

le gouvernement actuel- ou le prochain -pourra se prévaloir d'un succès s'il aura contribué à l'instauration d'une taxe sur les transactions financières.

d'une vraie taxe sur les transactions financières, une vraie TTF, qui rapporterait, monsieur le ministre, 57 milliards d'euros par an et permettrait de rembourser le plan de relance européen de 750 milliards d'euros, tout en finançant les dépenses de santé

avec un triple objectif : faire contribuer le secteur financier au redressement des finances publiques, exercer une action de régulation sur les marchés financiers et initier un mouvement d'adhésion des autres États au projet européen de taxation de la Commission. La TTF, conçue pour corriger l'ampleur des inégalités dues à la mondialisation, doit ainsi permettre au secteur financier de contribuer à la lutte contre les inégalités sociales croissantes. Ce besoin est plus que jamais d'actualité, exacerbé par les inégalités creusées par la crise sanitaire. Une augmentation du taux de 0,3 % à 0,5 % dégagerait 1 milliard d'euros de recettes supplémentaires.

Vous voyez bien qu'il y a un problème, qui traverse beaucoup de choix politiques de la France au sein de l'Union européenne. Le monde de la finance a été déconnecté des demandes de financement.

-venant élargir l'application de la procédure d'abus de droit dans certains cas où le contribuable a suivi les instructions ou circulaires émanant de l'administration fiscale. Antérieurement, il était établi que le principe d'opposabilité de la doctrine administrative faisait toujours échec à l'application de la procédure d'abus de droit, ce au titre du principe de sécurité juridique. Le Conseil d'État est revenu sur cette jurisprudence constante à la suite de la légalisation de la procédure de l'abus de droit par fraude à la loi, opérée par la loi de finances rectificative pour 2008. Il résulte pourtant des conclusions du rapporteur public que la volonté du législateur ne pouvait être identifiée en ce sens. Par ce revirement de jurisprudence, le Conseil d'État prive en partie le contribuable de la garantie législative d'opposabilité de la doctrine administrative, venant ainsi mettre à mal la sécurité juridique du contribuable qui se conformerait aux dires de l'administration, notamment, et surtout, en ce qu'il se verrait appliquer des majorations en sus de l'imposition rectifiée et des intérêts de retard. Ce dispositif aurait un coût budgétaire extrêmement limité, voire nul. De surcroît, il permettrait d'éviter toute application massive d'une erreur d'interprétation de l'administration,

entraîne une application automatique de la majoration de 80 %, ramenée à 40 % lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale des actes constitutifs de l'abus de droit ou qu'il en est le principal bénéficiaire, ce qui n'est pas le cas à l'article L. 64 B du livre des procédures fiscales, que vous citez. Il y a donc, me semble-t-il, une difficulté d'ordre technique. Par ailleurs, la décision du Conseil d'État que vous évoquez me paraît claire. Il y a effectivement dans notre droit ce que l'on appelle une garantie contre les changements de doctrine, laquelle permet au contribuable de se prévaloir d'une interprétation administrative. La garantie figure d'ailleurs à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. La loi protège alors le contribuable des changements d'interprétation par l'administration des textes fiscaux. Le Conseil d'État a simplement précisé que le contribuable ne pourra pas se prévaloir de cette garantie dans le cadre d'une procédure pour abus de droit s'il a eu recours à des montages artificiels à seule fin d'échapper à l'impôt. Cette décision ne remet pas en cause de manière générale la garantie contre le changement de doctrine. C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable.

qu'il a eu recours à un montage artificiel pour se prévaloir d'une doctrine et, en réalité, chercher à éluder l'impôt. La jurisprudence qui est ainsi posée nous convient

précurseur dans la réglementation du secteur de la et des crypto-actifs. Il a été conçu dans la concertation et fait consensus auprès de l'ensemble des acteurs, privés ou institutionnels. Ce dispositif souple avait vocation à élaborer une liste blanche la plus fournie possible, qui garantisse la protection des consommateurs. Tout son intérêt repose donc sur son attractivité pour les entreprises, qui sont invitées en nombre à entrer dans ce cadre légal. Pourtant, à ce jour, encore très peu d'entre elles ont obtenu une certification de l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour leur activité dans le domaine de la et des actifs numériques. Si la mise en place d'une contribution financière pour les acteurs bénéficiant des services de l'AMF semble légitime et juste au regard d'autres secteurs d'activité, instaurer une barrière à l'entrée pourrait toutefois remettre en cause l'utilité du dispositif, notamment lorsqu'il est optionnel. En outre, bien que dynamique, l'écosystème français de la reste de taille limitée. Aussi, le présent amendement a pour objet d'aménager ce dispositif de contribution, d'une part, en prévoyant que les émetteurs d'une offre au public de jetons et les prestataires de services sur actifs numériques aient

Cet amendement vise, dans le cadre des nouvelles contributions à l'AMF des acteurs de l'univers des crypto-actifs, à abaisser à la fois les planchers et les plafonds des montants pouvant être fixés par décret, tout en offrant un délai de six mois

pour s'acquitter de la cotisation. M. Rambaud a rappelé, à juste titre, que cela avait fait l'objet de l'un des articles de la loi Pacte. Il est, me semble-t-il, juste que ces nouveaux acteurs acquittent une contribution à l'AMF pour frais de contrôle, mais il faut veiller à ce qu'elle reste proportionnée

le mécanisme auquel notre commission des finances s'était fermement opposée lors de son instauration. En effet, le Sénat avait appelé le Gouvernement à substituer à ce que l'on avait qualifié d'artifice budgétaire

dans le cadre d'une convention signée entre l'Association française de la gestion financière et l'Autorité des marchés financiers, les sociétés de gestion ont accepté de financer de financer « volontairement » le nouveau référentiel centralisé des données du secteur, appelé « BIO-3 », pour un montant de 6 millions d'euros par an pendant cinq ans, soit 30 millions d'euros. Ainsi que nous l'avions craint ou anticipé, lesdites sociétés de gestion ont obtenu en contrepartie une baisse de leurs cotisations légales, mise en oeuvre par décret. Mes chers collègues, la Cour des comptes a, sans surprise, suivi la commission des finances en demandant la suppression de ce mécanisme en 2018.

Comme l'a dit M. le rapporteur général, c'est un point de divergence entre le Gouvernement et la commission des finances du Sénat. Nous considérons que l'article n'est pas un moyen de contourner le plafond des taxes affectées à l'AMF. D'ailleurs, cet article prévoit son rehaussement de 2,5 millions d'euros. Selon nous, il n'y a pas de menace sur l'indépendance de l'AMF, qui est construite sur un principe de séparation organique entre la commission des sanctions et le collège, qui est l'entité concernée dans la négociation de sa contribution. Par ailleurs, dans le contexte du Brexit, notre crédibilité passe aussi par la souplesse donnée par cet article. Nous sommes défavorables à la suppression

de bénéficier aussi du report en pied de facture du surcoût engendré par la disparition de la fiscalité avantageuse sur le gazole non routier (GNR). Ce secteur est tout prêt à se transformer, et notamment à acquérir des véhicules propres, mais, aujourd'hui, on en est plutôt à la phase d'expérimentation, et il faudra, demain, répondre à des problématiques, qui sont, d'une part, le surcoût de ces véhicules, ainsi que la plus faible autonomie frigorifique des solutions alternatives au GNR,

Je suis sûr que tous, ici, vous appréciez les huîtres et, si vous voulez en avoir pour égayer les fêtes à venir, si tant est que l'on puisse effectivement en profiter, il est nécessaire que des producteurs puissent proposer ces excellents produits. Les paysans de la mer,

La demande de retrait exprimée lundi ne portait pas sur la question de l'année d'imputation, à savoir 2020 ou 2021. Elle était liée au fait que, dans le cadre du plan de relance, nous prévoyons une enveloppe de 21 millions d'euros pour le secteur de l'aquaculture et de la conchyliculture.

celui-ci a suscité de nombreux amendements, ce qui prouve les inquiétudes et les interrogations de l'ensemble de nos collègues.

on relève une diminution des variables d'ajustement de l'ordre de 50 millions d'euros. D'un côté 26,7 milliards d'euros, et, de l'autre,

part, l'évolution de la population, pour la question de la dotation forfaitaire, d'autre part, le fait qu'il puisse y avoir un écrêtement forfaitaire dans le cadre du financement des variables d'ajustement, et, enfin,

en considérant que c'est effectivement, dans le contexte des finances publiques que l'on connaît, un premier effort. Je saisis l'occasion de l'intervention de M. Savoldelli sur l'évolution de la dotation de certaines communes du fait de l'évolution de leur éligibilité aux différents fonds de péréquation pour dire que, conformément à l'engagement que j'avais pris devant vous l'année dernière, vous trouverez à l'article 58 le mécanisme qui garantit la neutralisation des effets de l'évolution du panier de recettes fiscales des collectivités dans le cadre de la réforme de la taxe vous avez été nombreux à souligner, avec raison, que l'évolution du panier de recettes fiscales aurait des conséquences mécaniques, à recettes égales, sur le PFIA des collectivités, et que, donc, des difficultés se poseraient, comme en 2018, sur l'accès aux ressources de péréquation. Nous l'avons intégré à l'article 58, après des travaux avec le Comité des finances locales (CFL), et nous avons introduit le même mécanisme pour tenir compte des modifications de fiscalité locale que nous proposons, avec la diminution des impôts de production, de manière que ces deux réformes - TH et impôts de production -n'aient pas de conséquences sur le PFIA, et que cela ne modifie pas l'accès, ou plus exactement l'éligibilité ou la non-éligibilité, aux dotations de péréquation que sont la DSU et la DSR. C'est un engagement qui avait été pris et que vous retrouverez tenu à l'article 58. La parole est

-vous avez voté une dégradation des comptes publics, mes chers collègues : un petit 10 milliards d'euros avec la disparition des impôts de production pour l'année prochaine, et, comme

Cela dit, monsieur le ministre, vous avez tenté de nous rassurer en nous disant que vous aviez prévu le mécanisme qui permettrait de régler le problème que va poser la disparition de la taxe d'habitation.

vos propos rassurants valent peut-être pour l'exercice 2021, qui est l'année de basculement, sans encore de conséquences véritables sur des allocations de péréquation, mais de la suite ? ? Je le redis, comme je l'avais dit en discussion générale, les élus locaux ont aussi besoin de visibilité sur leurs dotations. Il y a déjà l'incertitude du post-2022 - on verra bien ce qu'il en sera -, mais il y a aussi cette inquiétude chez tous ceux qui bénéficient de la péréquation

aussi des conséquences positives en matière de neutralisation pour les années suivantes. Je précise également que le dispositif intégré à l'article 58 est exactement celui sur lequel nous avons échangé avec les membres du Comité des finances locales, et nous aurons de nouveau l'occasion, si c'est nécessaire, et autant que nécessaire, de les saisir pour continuer le travail.

en actes ; il est donc urgent d'augmenter le soutien financier de l'État aux collectivités, pour leur permettre de financer les postes d'ingénierie et d'animation territoriale nécessaires à la mise en oeuvre efficace de ces projets de relance et de transition écologique et sociale. En conséquence, cet amendement vise à augmenter la DGF.

afin de permettre aux collectivités territoriales et en particulier aux communes rurales de se doter de moyens supplémentaires en ingénierie, indispensables pour mener les investissements prévus dans le cadre du plan de relance. Nous le savons, nombreuses sont les collectivités territoriales qui connaissent une carence en matière d'ingénierie de projet, en dépit des besoins accrus qui se font ressentir sur les territoires. Les débats portant sur la création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ont illustré la nécessité de soutenir les collectivités qui devront accompagner la transformation des modes de production et de consommation, ainsi que le développement de l'économie locale, de l'emploi, ou encore de la transition écologique. Tel est l'objet du présent amendement. Son adoption permettrait de s'assurer que les crédits du plan de relance, dont il a été annoncé que l'exécution serait territorialisée, pourront réellement être consommés.

d'être à la croisée des chemins : nous devons prendre des décisions fortes pour continuer à nous engager réellement, sûrement, pleinement dans cette transition. Rien ne sera possible sans l'implication des collectivités territoriales. Nous devons donc leur donner les moyens de mettre en oeuvre ces grands changements, en leur faisant confiance, en faisant confiance à leur créativité, à leur inventivité, à leur connaissance fine des territoires, selon le principe de l'intelligence collective : on est meilleurs quand on est plus nombreux. Les élus sont des personnes engagées et impliquées. C'est pourquoi cet amendement vise à augmenter les moyens de fonctionnement des collectivités territoriales au service de la transition écologique, au travers d'une hausse de 700 millions d'euros de la DGF. L'amendement n° I-940, présenté

l'élaboration et la mise en oeuvre des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) sont obligatoires à l'échelle des intercommunalités de plus de 20 000 habitants. L'État a malheureusement toujours refusé de mettre en place un transfert de ressources pour que les intercommunalités puissent assumer cette nouvelle compétence obligatoire.

l'initiative de Jean-François Husson, le Sénat propose un mécanisme de contractualisation entre l'État et les intercommunalités, mécanisme fondé sur l'adoption du PCAET et le fléchage d'une partie de la contribution climat-énergie (CCE) vers le bloc communal. Nous proposions une contractualisation : vous adoptez un PCAET, vous recevez

elles ne peuvent être fléchées spécifiquement vers des dépenses dites « de transition écologique » ; prétendre le contraire serait méconnaître le principe d'autonomie financière de nos collectivités.

sein des villes et des départements concernés. Les gens qui font ces gestes de solidarité, d'accompagnement et d'aide alimentaire aux côtés des services publics communaux

Ce mécanisme avait été instauré pour garantir le respect de la trajectoire des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales.

n'est pas comme s'ils n'étaient pas plus affectés que l'État par la crise sanitaire ! Cela semble difficilement justifiable, pour ne pas dire inacceptable, dans un contexte où la trajectoire des concours financiers est devenue largement caduque. Dans le dispositif retenu par l'Assemblée nationale, cet article a également pour effet de reconduire en 2021 le plafonnement du prélèvement sur recettes

Aussi, dans l'attente d'une nouvelle définition de la trajectoire des concours financiers et des mécanismes permettant d'assurer son respect, cet amendement objet de ne pas adopter les nouvelles minorations de variables d'ajustement pour 2021 et de revenir sur le plafonnement sur recettes de la compensation de la réforme du versement transport.

sur l'engagement de l'État de compenser la perte de versement mobilité subie par les AOM. Il induit une baisse de recettes pour celles-ci, alors même qu'elles sont déjà confrontées à des pertes importantes du fait de la crise sanitaire. Il pénalise de surcroît les collectivités qui ont fait des efforts pour encourager l'installation d'entreprises et la création d'emplois. L'amendement

il n'est pas impossible d'inviter le Gouvernement à aller plus loin, notamment pour deux prélèvements qui sont aujourd'hui soumis aux variables d'ajustement et minorés à hauteur de 50 millions d'euros. Pour rappel, l'article 22 minore ce concours de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle à hauteur de 25 millions d'euros ; la dotation de transfert des compensations d'exonération de taxe d'habitation est également demandons donc que ces mesures injustes et difficilement acceptables pour les régions et les départements soient annulées.

les variables d'ajustement, parce que nous partageons les critiques qui ont été émises envers cet outil de régulation et de maîtrise de la trajectoire des concours de l'État aux collectivités. Cela m'amène à émettre un avis défavorable

La commande publique est en baisse de 22 % par rapport à 2019. L'Observatoire français des conjonctures économiques explique ainsi que la chute de l'investissement public au cours du premier semestre de 2020 est quatre à cinq fois plus forte que les retournements les plus sévères observés depuis 1950. L'horizon incertain des collectivités sur leurs finances risque d'amplifier cette tendance. Sans aides de l'État venant compenser leurs pertes de recettes et hausses de dépenses ni certitudes sur la fin de l'épidémie, les collectivités sont contraintes de réduire leurs dépenses plutôt que de creuser les déficits. Comme nous l'avons proposé dans notre proposition de loi de soutien financier aux collectivités, nous défendons l'introduction d'une clause de non-régression de la dotation globale de fonctionnement.

tout aussi bien le défaire ! La rédaction de cet amendement ne permet pas non plus une stabilisation à périmètre constant et courant du montant de la DGF

élu local » (DPEL) est attribuée aux communes dont la population prise en compte pour la DGF est inférieure à 1 000 habitants et dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants. Cette dotation est destinée à compenser certaines dépenses obligatoires entraînées par les dispositions législatives relatives aux autorisations d'absence, aux frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints. en somme de soutenir l'exercice par les élus de leur mandat dans les communes de petite taille. Or force est de constater que, dans les petites communes, la moindre variation de potentiel fiscal et financier peut avoir de lourdes incidences.

tout critère de richesse fiscale pour les communes, raison pour laquelle la commission sollicite son retrait.

à M. le rapporteur général. Les nombreux amendements qui vont être présentés témoignent de notre souci commun de soutenir les collectivités territoriales, dont la situation financière est fortement fragilisée par la crise. Nous sommes en droit de nous étonner que le Gouvernement ne propose aucune mesure de compensation financière en faveur du bloc communal et des départements pour l'année prochaine. Je rappelle que, contrairement à l'État, les collectivités n'ont pas la possibilité de s'endetter massivement. Il me semble donc que le Sénat joue pleinement son rôle en s'efforçant de combler cette lacune. Je vais vous exposer maintenant la position d'ensemble de la commission sur ces différents amendements qui, vous vous en doutez, ne pourront pas tous être adoptés. Tout d'abord, la commission a entendu assurer une compensation de l'intégralité des pertes de CVAE que subiront les communes, les EPCI et les départements en 2021, en comparaison de l'année 2020. Cette mesure, dont le coût pour l'État pourrait s'élever à près de 1 milliard d'euros, constitue donc un soutien financier massif en faveur des collectivités territoriales.

J'indique que la commission propose de supprimer l'article 22, afin de permettre aux collectivités de bénéficier pleinement de la dynamique de la TVA qui leur a été attribuée dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation, l'an passé. Cela représente un gain de 1 milliard d'euros pour les départements et de 300 millions d'euros pour les EPCI, par rapport au texte qui nous a été transmis par l'Assemblée nationale.

Malgré les propositions de notre collègue député Jean-René Cazeneuve en ce sens, le Gouvernement n'a pas fait ce choix. Nous le regrettons ! Ce mécanisme permettrait pourtant d'assurer un filet de sécurité garantissant une certaine visibilité des collectivités collectivités sur leurs ressources, et présenterait l'avantage de s'ajuster automatiquement à la perte réelle. Ces amendements contiennent deux améliorations du dispositif : d'une part, la prise en compte de la seconde période de confinement dans le calcul des pertes de recettes domaniales en 2020, et, d'autre part, l'intégration des régies communales et intercommunales dans son champ. En effet, dernières ne sont en principe pas éligibles au chômage partiel et n'ont fait l'objet d'aucune mesure de soutien. Le paquet de mesures que la commission vous propose d'adopter s'avère extrêmement favorable aux collectivités territoriales et représente déjà un effort financier pour l'État de

Le coût pour l'État d'une telle mesure serait, au demeurant, extrêmement élevé, exception faite du cas particulier de la compensation de la CVAE proposée à l'amendement de la commission et que l'État prévoit déjà, monsieur le ministre, pour les régions. La commission n'est pas non plus favorable aux amendements visant à compenser l'intégralité des pertes et des recettes tarifaires des collectivités, hormis, je le rappelle, le cas particulier des régies dont il a été question. En effet, une telle proposition pose des difficultés techniques qu'il n'est pas aisé de surmonter, en ce que cela impliquerait la prise en compte de choix de gestion très variables entre les collectivités territoriales, qu'il faudrait pouvoir neutraliser. Ainsi, la commission, conformément à sa position constante, est défavorable aux amendements qui entendent compenser les hausses de dépenses des collectivités territoriales. Eu égard aux autres mesures prises et proposées en faveur des départements,

: jamais, dans aucune crise traversée par les collectivités locales, l'État n'avait mis en place un mécanisme de garantie de recettes sur les recettes fiscales et domaniales. Cela vient s'ajouter à la stabilité globale des dotations

je pense notamment aux charges de personnels, qui ont pesé très lourdement sur les communes -afin, bien sûr, d'assurer la protection des citoyens et le maintien de nos services. Nous savons déjà que certaines recettes, telles que la CVAE, sont versées de manière décalée dans le temps, et que d'autres recettes ne reprendront pas aussi vite leur niveau d'avant-crise, par exemple la taxe de séjour. Les estimations de pertes de recettes seulement fiscales déjà constatées prévoient, pour l'année 2021, une baisse de 840 millions pour le bloc communal, de 560 millions d'euros pour les départements, et de 1,2 milliard d'euros pour les régions. Ces conséquences, amenées à évoluer, s'inscrivent bien, malheureusement, dans la durée. Nous souhaitons donc que ces conditions ne pèsent pas davantage

des hausses de dépenses des collectivités liées à l'épidémie de covid-19, sans distinction entre les différents échelons. Les six

Tel que prévu, le calcul du montant des pertes se fonde, non pas sur une comparaison avec l'année 2019, mais bien sur la moyenne des années 2017, 2018 et 2019, réduite du montant des évolutions d'autres recettes fiscales locales. Il ne comptabilise pas non plus les baisses de recettes tarifaires ni les dépenses engagées pour faire face à la crise. N'étant pas

Je propose donc la mise en place d'un dispositif qui permette de compenser réellement la perte de recettes. Il est prévu également de réparer une inégalité entre les communes qui ont décidé de gérer directement

nous n'avions pas traité la question des pertes de recettes tarifaires. Pour certaines communes, les pertes de recettes liées à l'occupation du domaine public sont importantes, alors que les recettes tarifaires ne le sont pas. Pour d'autres communes, c'est l'inverse.

permettront aux communes et aux EPCI à fiscalité propre de disposer d'une visibilité sur leurs ressources minimales en 2021, pour ainsi investir et participer à la relance. Ces collectivités seront confrontées, tout comme en 2020, à des pertes de recettes fiscales et domaniales. Ce sera aussi le cas pour les régies municipales dotées de la seule autonomie financière

dans les forêts de remplacement, où les communes forestières sont toujours mises devant des réalités financières qui ne leur permettent pas de boucler réellement leur budget. Je souhaiterais donc bien mettre l'accent sur les attaques de scolytes, qui sont reparties avec les températures clémentes du printemps, et sur la sécheresse actuelle, qui achève d'affaiblir les peuplements, de plus en plus dépérissants, dans nos forêts. L'avenir de certains massifs forestiers est clairement remis en cause. Épicéas, hêtres, frênes et chênes sont aujourd'hui victimes de toutes sortes de chenilles ou insectes qui pullulent.

et par la difficulté de réinvestir dans leurs massifs forestiers. Cet amendement vise à permettre la compensation des pertes de recettes liées à l'exploitation de la forêt.

départements et pour le bloc communal en 2021, avec un nouveau prélèvement sur recettes garanti sur l'année 2020. Il s'agit donc d'un ajustement automatique à la perte réelle

face à une crise d'une ampleur exceptionnelle. Le RSA était déjà un sujet de préoccupations. Depuis 2010, les dépenses de solidarité ont fortement augmenté avec le nombre d'allocataires.

ne cessent d'augmenter, et l'on n'arrive pas à obtenir la compensation pleine et entière à l'euro près de cette dépense des départements.